chers collègues, par lettre en date du mercredi 5 juin 2019, le Gouvernement a demandé l'inscription de la suite du projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé à l'ordre du jour du vendredi 7 juin, le matin, l'après-midi et, éventuellement, le soir. soir. Acte est donné de cette demande. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé

conformément au principe de pertinence des soins, vers les établissements de santé de recours et de référence ou vers les autres structures adaptées à leurs besoins telle rédaction laisse entendre que les hôpitaux de proximité seront avant tout des établissements qui orientent les patients vers d'autres structures de soins, notamment les hôpitaux généraux. Selon nous, l'hôpital de proximité doit d'abord être une structure d'accueil qui délivre des soins avec le souci d'assurer un meilleur maillage territorial du service public hospitalier. Je vous rappelle que, à l'automne dernier, lors de l'examen du budget de la sécurité sociale, le député En Marche Olivier Véran, a fait adopter un amendement expérimentant une incitation financière pour que les services d'urgences réorientent les patients vers les soins de ville dans la mesure du possible. Nous avons vraiment l'impression que les solutions du Gouvernement à la crise de nos hôpitaux, à force de proposer des panneaux de redirection, vont nous mener dans l'impasse.

Cet amendement vise à modifier la rédaction concernant la mission de permanence et de continuité des soins, pour souligner son caractère articulé et complémentaire avec les organisations mises en place sur les territoires. Ainsi, nous proposons de repositionner cette exigence au sein des missions partagées des hôpitaux de proximité avec les autres acteurs de santé du territoire. Il est en effet essentiel que la contribution des hôpitaux de proximité sur ces sujets se fasse en cohérence avec les projets des communautés professionnelles territoriales de santé. L'amendement vise par ailleurs à étendre la responsabilité territoriale partagée à l'ensemble des missions partagées et non pas uniquement à la permanence des soins, hôpitaux de proximité et professionnels de ville devant agir ensemble en faveur de l'état de santé de la population.

au service d'une population du territoire. Si le présent article 8 précise bien le cadre d'intervention global de ces établissements, il ne fait pas mention explicitement du rôle majeur que pourront avoir les hôpitaux de proximité en matière de continuité et de permanence des soins, en complémentarité de l'offre libérale, sur les territoires. Le présent amendement vise donc à préciser ces deux missions, considérées comme fondamentales par les usagers des services hospitaliers sur les territoires. Par ailleurs, alors que le présent projet de loi consacre la notion de télésoins en complémentarité des actes de télémédecine, il n'est pas fait mention du rôle majeur que pourront avoir les hôpitaux de proximité en matière de télésanté. Ceux-ci doivent pouvoir être de véritables plateaux techniques pour la réalisation d'actes de télésanté, utilisables par tous les professionnels de santé du territoire. Par cet amendement, il s'agit donc d'intégrer la télésanté comme mission pleine et entière des hôpitaux de proximité. Les

Amiel. Les hôpitaux de proximité doivent assurer la continuité et la permanence des soins. Pourquoi ces deux notions doivent-elles faire partie de leur mission ? Parce qu'il s'agit de proposer, quand c'est possible pour le patient, une première offre de soins pour tous les territoires et à tout moment. Nous n'opposons pas gradation des soins et permanence des soins, nous croyons que les deux notions fonctionnent ensemble. En effet, c'est justement la gradation qui permet de proposer une offre de soins de premier recours au plus près des populations.

Par conséquent, afin d'assurer la cohérence de cette première offre de soins, nous souhaitons voir la permanence et la continuité figurer au rang des missions des hôpitaux de proximité.

en sens inverse, pour que la prise en charge des patients se fasse au plus près de leurs besoins en proximité, dès lors que cela est compatible avec l'exigence de sécurité et la qualité des soins. Une série d'amendements vise à préciser dans les missions de l'hôpital de proximité leur contribution à la permanence des soins et au développement de la télésanté. Sur le premier aspect, la rédaction adoptée en commission a permis de mettre en exergue la contribution indispensable des hôpitaux de proximité à la permanence des soins et à la continuité de la prise en charge, en complémentarité avec les professionnels de ville. L'amendement n° 667 rectifié de Mme Guillotin me paraît le plus adapté il précise la rédaction adoptée en commission, tout en inscrivant plus explicitement cette exigence dans les missions des hôpitaux de proximité. La commission a donc émis un avis favorable sur l'amendement n°

d'hôpitaux aux missions différentes, vous êtes en train de porter un coup extrêmement important à notre système de santé publique, en affaiblissant davantage ce qui en fait la colonne vertébrale, à savoir l'hôpital public. En réalité,

quand les remèdes n'ont pas d'effets, on les change ! Mais on les change de fond en comble, ce que vous refusez de faire.

n'auront pas envie d'aller travailler dans ce genre de structures. Personnellement, je suis convaincu du contraire, puisque, dans les zones rurales défavorisées en matière d'équipement, elles constitueront une aide considérable à leur mode d'exercice.

en proximité. Si vous avez une infection urinaire haute, une pyélonéphrite, et que vous avez besoin d'antibiotiques intraveineux, vous serez hospitalisée dans un hôpital de proximité, vous n'aurez pas besoin d'un hôpital de recours. Même chose pour l'exploration d'une fièvre. Cette organisation,

induit un doute- je ne sais pas si je me fais bien comprendre ... Il semble en effet inutile de rappeler ce principe de gradation dans les pratiques, puisqu'il s'impose à tous les professionnels du soin. du soin. Si nous sommes favorables au développement de la gradation dans l'organisation et la mise en place du réseau des hôpitaux de proximité, nous estimons que la

Ainsi, le Haut Conseil s'est exprimé pour le développement « des établissements de santé communautaires assurant une ligne d'hospitalisation de premier recours, au service des médecins de ville, bien intégrés dans leur environnement, principalement axés sur la médecine polyvalente et la filière gériatrique, pouvant servir de point d'appui à la régulation des soins non programmés et des urgences, avec le cas échéant un plateau d'imagerie de proximité et de biologie de routine, et pouvant comporter, en fonction des spécificités territoriales, un centre de suivi de grossesse de proximité À partir de cette définition, nous proposons que les hôpitaux de proximité assurent bien une ligne d'hospitalisation de premier recours au service des médecins de ville, exercent une activité de médecine polyvalente comprenant des activités interventionnelles de jour et développent une filière de gériatrie. Ce à quoi il convient d'ajouter les consultations avancées et la prévention, notamment en addictologie. Madame la ministre, cette définition permettrait une clarification indispensable du rôle et des missions des hôpitaux de proximité comme premier niveau de la gradation des soins hospitaliers, susceptible d'encadrer l'ordonnance à venir, de manière à ce que le Parlement ne donne pas un blanc-seing à l'exécutif sur un sujet majeur pour l'avenir de notre système de santé et pour l'accès aux soins, question prégnante pour nos concitoyens. Quel commission ? Les précisions apportées par M. Jomier dans son amendement ne bouleversent pas l'équilibre des missions des hôpitaux de proximité. Elles paraissent même pertinentes, quoique déjà incluses dans le champ plus large esquissé par le texte. Il n'est sans doute pas utile d'énumérer dans la loi toutes les déclinaisons techniques et médicales des missions générales ici visées. Cet amendement me donne d'ailleurs l'occasion de demander l'avis du Gouvernement sur le contour des missions futures des hôpitaux de proximité, au regard des propositions faites par le Hcaam.

la notion d'« actes techniques » mentionnée à l'alinéa 7 que vous souhaitez amender recouvre notamment les activités interventionnelles. Ainsi, les hôpitaux de proximité, dans la rédaction actuelle qui vous est proposée, pourront pratiquer de telles activités dès lors qu'ils respecteront les conditions d'implantation et les techniques de fonctionnement de ces dernières. Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à cet amendement. La parole est à M. Bernard Jomier,

C'est volontairement que nous ne listons pas la totalité des spécialités. Pourquoi ? Parce que nous passons notre temps à dire que chaque territoire a ses spécificités. Oui ! Il est évident qu'un hôpital de proximité en banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis par exemple, aura besoin de déployer des activités spécifiques à

Comme l'a rappelé notre collègue Guillaume Arnell lors de la discussion générale, la fermeture de services de maternité dans certaines zones rurales risque d'aggraver la désertification médicale et d'accentuer l'absence d'attractivité de ces territoires, qui sont de plus en plus isolés. Les maternités et, tout particulièrement, les services d'obstétrique doivent former un maillage serré sur le territoire.

possible d'avoir partout un plateau technique de cardiologie ou de neurochirurgie. Nous devons être ambitieux : plutôt que de réduire les services en fonction des moyens et au gré de la détérioration des infrastructures, et donc de la sécurité des patients, nous proposons de définir les hôpitaux de proximité en fonction des besoins actuels et futurs. Comme l'a souligné ma collègue Laurence Cohen, nous proposons que chaque hôpital de proximité soit doté d'un service d'urgences ouvert en permanence. ouvert en permanence. Madame la ministre, vous allez certainement penser que je suis complètement obsédée par cette question, mais j'aimerais que vous puissiez m'assurer que, dans le Pas-de-Calais, à l'hôpital de Lens, le service d'urgences, qui est menacé, sera ouvert pendant les mois de juillet

de revaloriser les carrières et les rémunérations pour attirer les professionnels, d'améliorer les conditions de travail en recrutant des personnels soignants, des aides-soignants notamment, une excellence de proximité. L'excellence ne doit pas être réduite aux seuls services spécialisés, mais doit concerner l'ensemble de notre système de santé. Tels sont notre vision et notre projet. L'amendement

pour répondre au mieux aux besoins de la population et des bassins de vie. Cet amendement vise à ce que les hôpitaux de proximité puissent exercer une activité dite de petite chirurgie. En effet, il est essentiel que les hôpitaux de proximité soient en mesure de proposer une offre de santé la plus complète possible aux publics qu'ils couvrent. S'il n'apparaît pas réaliste de permettre à chaque hôpital de proximité de disposer d'un service de réanimation, en raison du faible nombre d'opérations, il est néanmoins capital qu'ils puissent pratiquer des actes de chirurgie ne nécessitant pas le recours aux techniques d'anesthésie générale. L'amendement

dont nous avons déjà parlé : quelles doivent être les missions des hôpitaux de proximité ? Ont-ils vocation à proposer l'ensemble des services hospitaliers ? J'entends tout à fait l'exigence de proximité dans l'accès aux soins

à l'échelle des territoires selon une logique de complémentarité. Il ne faut pas voir dans cette évolution qu'un risque de déclassement pour certains établissements : nous souhaitons aussi que des établissements de santé qui rendent un service de proximité puissent monter en gamme et soient consolidés dans leurs missions en devenant hôpitaux de proximité.

à ce que les 243 établissements qui relèvent aujourd'hui de ce statut le perdent demain, car nous savons bien que nous ne pouvons maintenir des plateaux techniques poussés, où seraient présents des anesthésistes en nombre suffisant, dans tous les établissements de santé. Il me semble que l'évolution que vous proposez se ferait en définitive au détriment d'un grand nombre d'établissements, qui perdraient un mode de financement plus adapté à leur rôle de service public de proximité. Les amendements n 774 rectifié et 775 rectifié sont en partie satisfaits,

l'amendement n° 614 rectifié, qui a été retiré, il était satisfait par le texte. Concernant l'amendement n° 719 rectifié, la commission considère qu'il appartiendra à la Haute Autorité de santé de déterminer quels sont les actes de chirurgie qui pourront être concernés par cette dérogation.

répondre le mieux possible, à l'aide des nouvelles techniques, aux besoins de la population. Mais, je le répète, plus d'hôpitaux de proximité, c'est moins d'hôpitaux généraux ! La parole est à Mme Céline Brulin,

d'ailleurs regretter que, année après année, les crédits en faveur de la prévention n'augmentent pas, voire diminuent. Mais, même si on met le paquet sur la prévention, ça ne remplacera pas nos hôpitaux de proximité

explication de vote. Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, ou Hcaam, a avancé des pistes dans un rapport remis au Premier ministre. instance a du mal à comprendre votre stratégie, madame la ministre ! Le rapport d'experts préconise de multiplier les petits hôpitaux de proximité. Toutefois, la dernière réforme a mis en place les groupements hospitaliers de territoire. Malheureusement, on fait tout le contraire,

Nous avons prévu que les SMUR, les services d'urgences ou des centres de périnatalité puissent être maintenus dans des hôpitaux de proximité, en fonction des besoins du territoire et de l'offre avoisinante. Bien entendu, si le premier service d'urgences est à 200 kilomètres, nous nous poserons la question du maintien d'un SMUR.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est ouvert.

la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

la lutte contre la désertification médicale. Il s'agit de répondre ainsi à une inquiétude profonde qui traverse nos territoires et de réaffirmer un principe qui a besoin d'être rappelé : la santé est aussi une affaire d'aménagement du territoire et de respect de l'égalité entre territoires.

des maternités, à des plateaux techniques hospitaliers et à des services d'urgences de proximité dans un rayon d'environ trente minutes autour de leur domicile. Une approche territoriale de la politique de santé permettra de lutter contre ce phénomène. Les hôpitaux de proximité peuvent représenter le fer de lance d'une lutte sanitaire salutaire et fondamentale pour les Français. Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter pour cet amendement, qui tend à faire de ces hôpitaux un outil de lutte

avec les acteurs de l'ambulatoire, pour être des catalyseurs de l'accès aux soins dans les territoires. Leur responsabilité territoriale, partagée avec les autres acteurs de santé, est déjà explicitement mentionnée. Quant

Merci,

Plutôt que de raisonner en termes de fermetures, et donc de concentration, ne serait-il pas possible de fonctionner en réseau, en déplaçant les professionnels, de manière à favoriser des services de qualité ? ce cas particulier, ce serait particulièrement facile, dans la mesure où la maternité la plus proche est située au sud d'Autun, à environ une vingtaine ou une trentaine de minutes, ce qui permettrait de maintenir deux sites et de disposer, du point

La médecine française s'est organisée autour de l'hôpital et des CHU. Dans ce schéma, la médecine générale ne semble pas être reconnue à sa juste valeur. Même s'ils ont une activité ambulatoire exclusive en ville et à la campagne, les généralistes sont principalement formés en milieu hospitalier. Les diplômés ont donc une vision erronée des territoires. L'accès aux soins pour tous, garanti par l'ordonnance du 4 octobre 1945, n'est aujourd'hui pas totalement assuré ; il demeure des zones sous-dotées en médecins généralistes,

pour répondre à ces enjeux ; cela passe par la facilitation de l'installation des médecins libéraux sur tout le territoire, en assurant une partie de leur formation dans des centres ambulatoires universitaires. Quel

L'article 8 du projet de loi ne prévoit, comme activité de soins socle obligatoirement assurée par l'hôpital de proximité, que la médecine. Ce faisant, il exclut toute possibilité, pour des établissements de santé, publics ou privés, qui n'assurent qu'une activité de soins de suite et de réadaptation d'obtenir la qualité d'hôpital de proximité. Cela revient donc à exclure, par principe, près de 150 cinquante établissements de santé, dont une grande partie assure pourtant une offre de soins et de prise en charge de proximité, en lien étroit avec les professionnels de santé de premier recours et de soins spécialisés. soins spécialisés. Ces établissements pourraient renforcer le maillage territorial des hôpitaux de proximité, spécialement dans les zones rurales ou éloignées des grandes agglomérations et des métropoles. C'est pourquoi le présent amendement a pour objet de permettre que des établissements de santé publics ou privés assurant aujourd'hui une activité de soins

Le projet de loi ne représente donc pas un recul en la matière par rapport à la situation actuelle. On peut comprendre que, pour assurer le premier niveau de la gradation des soins hospitaliers, les hôpitaux de proximité doivent proposer une activité de médecine. Il serait toutefois important que des établissements de SSR soient accompagnés,

certaines de ces structures pourraient organiser une forme de transition vers un hôpital de proximité. Ce qui compte, en réalité, ce sont les missions socles que nous donnons aux hôpitaux de proximité- la médecine, un plateau technique de radiologie et de biologie -, et,

plus d'un tiers des découvertes de séropositivité sont trop tardives. Ces chiffres sont dus, pour une large part, à un manque d'information, à un manque d'accès et à une stigmatisation encore trop présente. Dans cette perspective, le traitement post-exposition est un dispositif d'urgence qui doit être engagé le plus vite possible après exposition au risque, au mieux dans les quatre heures et au plus tard dans les quarante-huit heures. Afin de permettre aux personnes ayant été exposées à un risque de contamination de réagir au plus vite et de limiter de façon importante le risque de contamination par le virus, grâce au TPE, il apparaît essentiel que le maillage territorial des structures pouvant le prescrire soit le plus fin possible. Pour faire face à cette réalité, notre amendement vise à ce que les hôpitaux de proximité se dotent obligatoirement d'un dispositif spécialisé pour l'accueil et la prise en charge des victimes d'un accident d'exposition à un risque viral et puissent prescrire un traitement post-exposition. Quel

Aussi cet amendement vise-t-il à inclure dans les missions des hôpitaux de proximité le dépistage des maladies chroniques chez les patients à risques, notamment celles identifiées comme prioritaires dans la stratégie Ma santé 2022.

confier une mission générale de prévention et de promotion de la santé. Cela permet évidemment de viser des actions de dépistage des maladies chroniques chez les patients à risques sans qu'il soit besoin de les mentionner spécifiquement dans la loi. La commission demande donc le retrait de ces deux